La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Pourtant, le 7 janvier dernier, Lucas s'est donné la mort. Pourquoi, en 2023 en France, un gamin homosexuel en arrive-t-il à se suicider ? Parce que- et, croyez-moi, je sais trop bien de quoi je parle -, à n'envisager qu'une vie de moqueries, de rejet, d'exclusion et de haine, on en arrive parfois à ne plus envisager de vie du tout. C'est donc avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de gravité, que je voudrais m'adresser aujourd'hui à toutes celles et à tous ceux, y compris au Gouvernement, dont les propos ont nourri et nourrissent ces violences à toutes celles et à tous ceux qui ont marché avec La Manif pour tous, qui ont raconté que nos familles étaient contre-nature, que nos droits étaient d'égoïstes caprices, que respecter les mineurs trans, c'était de l'idéologie, qu'apprendre aux élèves le respect de la diversité, c'était de la propagande, que moi, j'étais un problème lorsque je publie des photos avec ma compagne, précisément pour donner à voir à des adolescents comme Lucas un avenir dans lequel ils peuvent avoir une place et- pourquoi pas ? -devenir un jour un élu de la République ; à toutes celles et à tous ceux qui, par homophobie, par transphobie, parfois par simple cynisme électoraliste, nous prennent pour des boucs émissaires. Si le suicide de jeunes LGBT vous peine, si vous voulez réellement que cela s'arrête, commencez par le commencement ! Faites votre examen de conscience ! Dites-nous que vous vous êtes trompés, que ce drame vous a fait comprendre quelque chose : que nous étions non pas une idéologie, un argument de campagne, mais des humains ? Lucas, Dinah, Luna auraient pu être vos enfants, vos petits-enfants. Et leurs harceleurs aussi. Les enfants entendent et répètent ce que les adultes racontent. L'école est dans la société. Elle est traversée par ses débats, nourrie par ses haines et pétrie par sa violence. Aurez-vous pour la famille de Lucas, pour ses amis, l'humilité de changer ?

le chagrin, la douleur. Il n'y a pas de mots ... Que voulez-vous que je vous dise ? J'adresse mes pensées les plus émues à ses parents, à ses proches, à ses amis. Ce drame montre à quel point la lutte contre le harcèlement scolaire, la lutte contre l'homophobie- parce que, oui, l'homophobie tue ! -doit demeurer une priorité du Gouvernement. L'orientation sexuelle est souvent un point d'appui des auteurs de harcèlement. C'est vrai aussi d'autres caractéristiques, comme l'apparence physique, l'origine, la condition sociale.

En matière d'homophobie et d'égalité entre les femmes et les hommes, la prévention passe en particulier par l'éducation à la sexualité. C'est pour cela que, dès le mois de septembre dernier, j'ai pris des mesures pour rendre effectifs ces enseignements, qui, admettons-le, ne sont pas correctement assurés aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir récemment avec les sénatrices Annick Billon,

Les larmes de sirène sont des granulés de plastique à usage industriel qui, à l'instant où je vous parle, viennent, poussées par des vents de l'ouest, envahir nos côtes et nos plages de Loire-Atlantique et de Vendée. moins visibles qu'une marée noire, mais si nombreuses et si petites qu'il est impossible de les ramasser toutes, malgré les efforts des associations et des collectivités territoriales. Je tiens à saluer ici l'arrivée du Centre de documentation, Les larmes de sirène se dégradent avec le temps en microparticules dans l'air et dans l'eau. Cette pollution est un véritable désastre pour la biodiversité. La contamination tue la vie marine. Les poissons ingurgitent toujours plus de plastique, qui se retrouve ensuite dans notre alimentation. Nous ingérons entre 39 000 et 52 000 particules de microplastique par an. C'est un enjeu de santé publique. La loi et des décrets obligent les entreprises à se doter d'équipements limitant la fuite de ces granulés et à mettre en place des mesures de protection. Cela n'apparaît plus suffisant, puisque la pollution actuelle provient du transport maritime. Une telle atteinte à l'environnement est inadmissible ; nous devons agir plus fortement. Nous n'avons aucun moyen de retracer précisément l'origine de cette pollution. Les containers perdus en mer ne sont pas déclarés ! Nous ignorons la provenance des navires, leur destination et, bien entendu, les quantités transportées L'Organisation maritime internationale est chargée de prévenir des pollutions. Que fait-elle en la matière ? Quelle suite sera donnée à la plainte contre X des maires de Pornic, Jean-Michel Brard, et des Sables-d'Olonne, Yannick Moreau ?

Le Président de la République l'a redit hier, nous accueillerons au printemps une session de négociations du traité international sur l'élimination des plastiques. Ce doit être l'occasion pour nous de pousser sur le sujet.

Ce projet ne pouvait pas être reporté. Il eût été irresponsable de ne pas débattre de la question, et nous avons l'intention de le faire. S'est invité dans ce débat

Madame la Première ministre, allez-vous vous résigner à un tel naufrage, qui compromettrait définitivement notre régime de retraite

Je pense en réalité que cette question s'est invitée depuis longtemps dans le débat sur les retraites. La principale explication au déficit que nous connaîtrons dans les prochaines années si nous ne faisons rien est précisément d'ordre démographique. Vous le savez comme moi,

non seulement de maintenir la possibilité de valider des trimestres au titre de la parentalité, mais aussi de prendre en compte les trimestres particuliers cotisés au titre de l'assurance vieillesse du parent au foyer dans les critères d'éligibilité au minimum de pension

D'autres pays européens doivent procéder à la livraison de blindés lourds. La Pologne attend le feu vert allemand pour faire de même. La France conforte son aide militaire et livrera prochainement à l'Ukraine des chars de combat légers AMX-10 RC nous ne pouvons que le saluer. Cependant, compte tenu de la gravité de la situation et du nombre d'Ukrainiens qui perdent la vie chaque jour, la France et l'ensemble des pays européens ne peuvent pas différer plus longtemps la livraison des matériels blindés encore plus performants qui servent aujourd'hui à l'entraînement de nos armées et que l'Ukraine réclame avec insistance. La livraison de chars lourds, de missiles et de lanceurs sol-air permettrait aux forces ukrainiennes de protéger davantage les civils et d'être équipées d'un matériel de qualité reconnue.

Monsieur le ministre, allez-vous compléter la livraison des chars AMX 10 RC par des chars Leclerc et de nouveaux systèmes antimissiles ?

D'autres cessions pourront être envisagées dans les temps qui viennent. On parle beaucoup des chars ce mois-ci ; au mois de décembre, on parlait beaucoup de la défense sol-air. Je rappelle que, sur le segment de défense sol-air, nous aurons des choses à proposer à l'Ukraine dans les prochaines semaines, notamment sur les couches les plus élevées de défense du territoire ukrainien. La parole est à M.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Madame la Première ministre, vous qualifiez votre projet de réforme des retraites de « juste », « solidaire » et « pérenne ». Telle n'est pourtant pas la réalité. Pourquoi ? Votre projet est injuste, puisque vous portez la durée de cotisation à quarante-trois annuités et l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ce sont principalement les ouvriers, les employés et les femmes qui seront pénalisés. Votre projet est injuste, puisque les salariés les mieux rémunérés vont davantage capitaliser pour leur retraite tandis que la grande majorité des travailleurs ne pourront pas bénéficier du minimum de pension à 1 200 euros brut. Votre projet est injuste, car vous allez appauvrir les seniors, qui seront plus longtemps au chômage et que vous avez précarisés à l'extrême. Votre projet ne sera pas pérenne, car vous ne changez pas le logiciel du financement. D'autres solutions existent pourtant : il suffirait, et ce n'est qu'un exemple, de taxer de 2 % la fortune des milliardaires. Vous avez versé 160 milliards d'euros aux entreprises, sans contrepartie, pendant la crise du covid-19. Ce « quoi qu'il en coûte » ne peut-il être décidé pour garantir une réelle retraite, en bonne santé, une retraite sereine ?

Des voix s'élèvent pour souligner l'inconstitutionnalité de votre démarche. Madame la Première ministre, c'est parce que cette réforme voulue par Emmanuel Macron est injuste et parce qu'elle frappe les plus faibles qu'elle est rejetée très massivement. Avec l'ensemble des syndicats, la société tout entière est vent debout contre votre projet. Seuls le Medef et M. Ciotti vous soutiennent encore. Madame la Première ministre, nous relayons ici le vaste mouvement qui s'enclenche. Dès demain, le 19 janvier, nous serons dans la rue, avec le peuple, qui exige le retrait de votre projet

comme vous, je suis profondément attachée à notre système de retraite par répartition. Comme vous, je considère que c'est l'un des piliers de notre modèle social. Et- j'en suis sûre -comme vous, je veux que les jeunes d'aujourd'hui aient une retraite demain. madame la sénatrice Assassi, nous sommes confrontés à des faits : le nombre d'actifs baisse par rapport au nombre de retraités. Ce n'est pas une opinion ; c'est un constat. Si nous ne faisions rien, nous creuserions inévitablement les déficits et nous serions conduits à baisser les pensions ou à augmenter les impôts, voire à remettre en cause notre système de retraite par répartition. Et cela, avec le Président de la République, nous n'en voulons pas C'est pourquoi j'ai présenté la semaine dernière notre projet pour l'avenir de nos retraites. C'est un projet d'équilibre : nous demandons aux Français qui le peuvent de travailler progressivement plus longtemps. Et je mesure ce que cela représente

d'aller au-delà des quarante-trois annuités de cotisation, mais c'est la condition pour préserver notre système de retraite par répartition.

un projet de justice. Nous allons ainsi améliorer le dispositif dit « carrière longue ». Celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d'un départ anticipé de deux ans à six ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Nous reconnaissons mieux la difficulté de certains métiers en prenant en compte de nouveaux facteurs d'usure professionnelle, en favorisant les départs anticipés pour raisons de santé, en prenant le tournant de la prévention et en facilitant les reconversions. Les personnes en invalidité, en incapacité ou en inaptitude pourront bénéficier d'une retraite à taux plein à 62 ans. Au total, Français sur dix, souvent les plus modestes, les plus fragiles, celles et ceux qui exercent des métiers difficiles, pourront partir avant 64 ans. Ce sont les 20 de travailleurs les plus modestes qui auront le moins à décaler leur départ à la retraite. Notre projet, madame la sénatrice, est aussi un projet de progrès social.

nous avons la responsabilité d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition, parce que c'est lui qui protège les plus modestes. C'est grâce à lui que nous assurerons par la solidarité nationale une retraite digne à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé toute leur vie. La parole

Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, je souhaite vous parler aujourd'hui de « Zibac ». Je veux vous rassurer, mes chers collègues, il ne s'agit pas d'un talent émergent sur la scène musicale rap parle bien du développement des zones industrielles bas-carbone (Zibac). Ce programme vise à accompagner les territoires industriels dans leur transformation écologique et énergétique pour gagner en compétitivité et en attractivité.

qui représentent à elles seules près de la moitié des émissions industrielles de CO2 en France. Elles recevront 17 millions d'euros pour concevoir de nouveaux modes de production et de captation du CO2. Je salue cette politique, qui vise à créer une synergie entre notre engagement pour le climat par une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030 et la réindustrialisation de notre territoire, pour assurer notre souveraineté énergétique, favoriser l'emploi, l'innovation, la formation et conforter notre attractivité. Pour le Dunkerquois, c'est une incroyable opportunité. Ce territoire, que l'on considérait voilà encore quelques années comme relégué économiquement, marqué à jamais par les conséquences économiques et sociales de la crise portuaire et sidérurgique, est aujourd'hui un modèle inspirant en matière de transition écologique, énergétique et économique. Grâce à cette nouvelle ambition industrielle, des laboratoires sont créés, scrutés et enviés pour leur dynamisme. L'espoir et la fierté sont de retour. Ce sont près de 16 000 emplois qui sont attendus sur le littoral dunkerquois dans les dix années à venir. Permettez au Nordiste que je suis d'en être plus que satisfait. Le travail est colossal, mais exaltant, le bassin en question représentant 21 % des émissions industrielles de CO2. Le site d'ArcelorMittal a déjà mis en place un processus de recyclage de l'acier, ce qui permet de réduire d'un million de tonnes les émissions annuelles de CO2. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser davantage les actions lancées dans ce cadre sur les sites retenus et leur lien avec le futur projet de loi pour l'industrie verte ? La parole est à M.

: le défi de l'industrie verte et de la décarbonation industrielle. Ce doit être l'occasion historique pour la France d'inverser la tendance, après trente années de délocalisations industrielles,

Nous en annoncerons une dizaine d'autres d'ici à quelques semaines sur la base des réponses à l'appel à projets qui a été lancé à la fin de l'année 2022. Ce dispositif se complète de deux autres actions stratégiques, que nous menons sous l'autorité de la Première ministre et du Président de la République. La première est d'avoir une énergie décarbonée au prix le plus faible possible. C'est ce qui justifie la relance du secteur nucléaire en France, qui est un atout absolument stratégique pour gagner cette bataille de l'industrie verte.

à la relance des qualifications, des formations et à la valorisation des métiers industriels. Nous voulons également réfléchir à la manière de réserver nos subventions et nos soutiens financiers à des productions productions réalisées en Europe, et non pas en Chine ou ailleurs. Bref, nous voulons faire de ce projet de loi pour l'industrie verte l'un des moteurs, avec les zones dont vous avez parlé, de cette réindustrialisation, qui permettra à la France de retrouver son rang de grande puissance industrielle.

Voilà près de deux ans, j'interrogeais déjà Mme Barbara Pompili sur l'explosion des factures énergétiques, qui impactait alors fortement nos concitoyens. Aujourd'hui, la crise énergétique est encore plus alarmante et difficilement supportable pour les particuliers, les collectivités, les agriculteurs et les entreprises. Alors que l'objectif initial du marché européen de l'énergie était de faire baisser les prix, le constat est une nouvelle fois le même : le libéralisme à outrance ne tient pas ses promesses. En 2021, les tarifs de l'électricité avaient déjà augmenté de 60 % depuis l'ouverture du marché en 2007, preuve que le conflit en Ukraine n'est pas la seule explication. Face à cette crise, les textes, nationaux et européens, passent les uns après les autres, mais ce ne sont que des rustines d'argent public qui financent allégrement les fournisseurs alternatifs et ne permettent pas de mettre un terme aux dysfonctionnements et errements du marché de l'énergie. Monsieur le ministre, des solutions sont pourtant proposées sur l'ensemble des travées de la chambre haute : elles doivent être enfin écoutées ! Alors qu'une proposition législative pour réformer le marché de l'énergie sera présentée par la Commission européenne dans les mois à venir, la France doit prendre toute sa part dans ces négociations, en n'évitant aucun sujet. La décorrélation entre les prix du gaz et ceux de l'électricité, le maintien de l'ensemble des tarifs réglementés de vente et leur rétablissement pour les collectivités, les hôpitaux, les petites et moyennes entreprises et les exploitations agricoles, ainsi que la préservation des concessions hydrauliques en dehors des logiques du marché, doivent être des priorités dans ces négociations. Comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, avec à la clé une baisse des factures d'électricité de 10 % à 20 %, la France doit également demander une dérogation temporaire pour fixer le prix de l'électricité en fonction de son propre mix énergétique. En ce sens, reprendre la main sur un tel marché nécessite d'avoir un opérateur historique avec de réelles capacités d'investissement.

et ils règlent déjà plus de la moitié de la facture grâce à la contribution sur la rente inframarginale que nous avons mise en place et qui va rapporter cette année 26 milliards d'euros.

ou 1 000 euros le mégawattheure ? Oui, bien sûr, et je recevrai la semaine prochaine les fournisseurs d'énergie pour les rappeler à leurs obligations. Je vous le dis, ces 280 euros le mégawattheure doivent être payés, au moins en partie, par les fournisseurs d'énergie.

que le prix de l'énergie en France soit fixé en fonction du coût de production, et non pas au coût marginal d'ouverture de la dernière centrale à gaz.

nous avons repris le contrôle de 100 % d'EDF, ce qui devrait vous réjouir. Nous estimons, comme vous, que l'énergie est un bien stratégique et que l'électricité sera la grande question économique du XXI siècle. En prenant le contrôle de la production d'électricité décarbonée en France, nous nous donnons tous les moyens d'être compétitifs et d'avoir une économie qui réussit.

Les atteintes graves ou maltraitances envers les résidents persistent, et certaines sont systémiques. Mme Claire Hédon propose ainsi plusieurs actions à mener d'urgence pour mettre fin à ces situations inacceptables et restaurer la confiance des résidents et de leurs familles. Je ne peux que souscrire à ces prescriptions. Et, bien modestement, j'en ajouterai une : le soutien au financement des Ehpad publics, car ces établissements cherchent non pas à faire du profit, mais simplement à rendre un service de qualité, tout en équilibrant leurs comptes. qui sont ancrés au coeur de nos territoires et de nos collectivités locales, connaissent actuellement une situation financière dégradée, avec une capacité d'autofinancement négative. Il y a plusieurs raisons à cela des taux d'évolution des tarifs, fixés en fin d'année 2021, avant l'annonce de la revalorisation du point d'indice des personnels et l'explosion de l'inflation, sans oublier le sous-financement des mesures pérennes, comme le complément de traitement indiciaire, les mesures d'attractivité du Ségur ou la revalorisation des carrières. Sans prise en considération de ces éléments, les Ehpad publics ne pourront pas continuer à exercer, laissant au seul secteur privé la responsabilité de l'accueil des personnes âgées. Voilà quelques jours, le maire de Frontignan, dans l'Hérault,

mettre à jour le plan Solidarité grand âge, qui date de 2006, en prenant en compte la situation des Ehpad publics ? La parole

des tarifs hébergement et dépendance. Il importe de concilier une réalité, qui est celle du juste financement de ces établissements, dont dépend la qualité de service et d'accompagnement des personnes âgées,

s'attaquer à des causes plus structurelles, dont l'attractivité des métiers, le recours à l'intérim, qui a aussi un coût très élevé, et les taux d'occupation, qui sont aujourd'hui trop

madame la ministre, mes chers collègues, chaque jour, nous sommes alertés par les élus locaux et par les artisans et commerçants de nos territoires sur la flambée des prix de l'énergie. Boulangers, bouchers, restaurateurs, hôteliers, acteurs du tourisme, de la montagne : tous sont touchés de plein fouet par cette crise inédite. Les TPE-PME du monde rural sont confrontées à une hausse de leurs charges d'autant plus importante qu'elles supportent aussi des coûts de transport très lourds. La situation dans nos départements devient très préoccupante Dernièrement, dans un communiqué de presse, l'Assemblée des départements de France a formulé plusieurs demandes. Elle a appelé à restaurer l'autonomie que la décentralisation avait conférée aux départements pour pouvoir répondre au besoin de proximité de nos concitoyens, mais également à sortir de la logique de dérégulation du marché de l'électricité. Ces propositions sont légitimes et bienvenues pour éviter les dépôts de bilan, les licenciements, tout simplement la disparition de la vie dans nos territoires par la fermeture des commerces de proximité.

Nous produisons une électricité à un prix peu élevé grâce à notre parc nucléaire et à notre hydroélectricité. Nous ne pouvons plus sacrifier notre tissu économique et social et mettre le pays tout entier en grave danger pour conserver « quoi qu'il en coûte » notre participation à un marché européen de l'électricité dérégulé. Celui-ci s'est retourné contre nous, ce qui nous pénalise fortement dans les circonstances actuelles. Le Gouvernement va-t-il enfin entendre cet appel pour la décorrélation du prix de notre électricité de celui du gaz ?

ce dispositif est essentiellement financé par la récupération des profits réalisés par les fournisseurs d'électricité, qui ont bénéficié d'une augmentation des prix n'ayant rien à voir avec le coût de revient de leur propre production ou avec leur coût de

nous travaillons à une réforme du marché permettant aux Français de bénéficier d'un prix de l'électricité qui représente la réalité de la production électrique française. Non ! Oui, la Commission européenne a évoqué à la fin de l'année 2022 un cadrage de cette réforme qui va dans le sens

Madame la ministre, tout cela est trop long. Venez dans nos territoires voir les entreprises qui sont en train de fermer. Il est urgent d'agir

collègues, au printemps 2021, je défendais avec le groupe socialiste une proposition de loi visant à imposer la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme ubérisés que Mme la Première ministre, alors ministre du travail, rejetait d'un revers de main. Depuis, la Commission européenne, sous l'impulsion de Nicolas Schmit, a présenté au mois de décembre 2021 une proposition de directive reprenant ce principe, et le Parlement européen adoptera une position en faveur de ce texte dans les prochains jours. Dans le même temps, vous ne parvenez pas, et c'est heureux, à convaincre les autres gouvernements de venir sur vos positions, comme en atteste l'isolement de la France au sein du Conseil des ministres de l'Union européenne. Monsieur le ministre du travail, alors que le Président de la République se fait le chantre de la construction européenne, alors que la majorité des institutions et de plus en plus de gouvernements se prononcent en faveur de la présomption de salariat, et donc d'une véritable avancée sociale à l'échelle européenne, quand allez-vous changer de position ?

Le droit français est connu : il a été fixé dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, qui a donné lieu à deux ordonnances, elles-mêmes ratifiées par le Parlement- en tout cas la première -, et qui fixent justement ces principes de représentation. Depuis, il y a eu l'initiative de la Commission européenne visant à faire adopter par le Parlement et par le Conseil une directive sur le droit des travailleurs de plateforme. Vous dites que la France est isolée

que les travaux pourraient aboutir à la fin de la présidence espagnole, c'est-à-dire à la fin du second semestre de 2023. Nous sommes convaincus de pouvoir trouver, dans le dialogue, une position qui soit respectueuse de chacune des législations nationales, tout en permettant de garantir le droit des travailleurs de plateforme. Dans l'attente, nous continuons à travailler à l'échelon national. À la fin du mois d'octobre dernier, j'ai installé les premiers groupes de travail à la suite des élections visant à désigner les représentants tant des plateformes que des travailleurs des plateformes. Le dialogue est fécond, puisque, dans quelques minutes, avec Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports, nous rejoindrons les locaux de l'Autorité des relations

nous permet de montrer à nos partenaires européens que nous pouvons concilier l'indépendance, l'entrepreneuriat et la protection des droits sociaux.

on ne passe pas facilement de l'enregistrement de 15 000 brevets par an à la gestion de 5 millions de formalités concernant les créations d'entreprises, les modifications et les cessations. Surtout, on ne simplifie pas en se contentant de numériser sans alléger les procédures. Sur l'année 2022, ce service a été marqué par de nombreux dysfonctionnements et blocages. Depuis le 1 janvier 2023, le site est la voie unique obligatoire pour effectuer les différentes formalités d'entreprise. Malheureusement, une attaque informatique l'a rendu inutilisable du 3 janvier au 7 janvier ! Monsieur le ministre, quand ce guichet unique fonctionnera-t-il correctement et, surtout, quand sera-t-il simplifié pour que nos entrepreneurs produisent de la valeur plutôt que des renseignements administratifs ?

à un seul, de 56 formulaires à un seul, et de 70 % de démarches écrites à 100 % de démarches numérisées. J'y insiste, c'est un facteur de simplification majeure. Est-ce que la situation actuelle est satisfaisante ? Non Non ! D'abord, nous avons été l'objet, comme vous l'avez rappelé, d'une cyberattaque, avec 120 000 connexions par seconde qui ont saturé le site. Il a fallu le remettre en état, ce qui nous a pris quelques jours. a pris quelques jours. Par ailleurs, sur l'ergonomie même du site, il reste des améliorations à apporter ; je le reconnais bien volontiers. Est-ce que nous faisons le nécessaire ? Oui ! Nous avons reçu hier le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, et nous lui avons demandé des corrections. nous lui avons demandé des corrections. Nous sommes à l'écoute de tous ceux qui créent leur entreprise ou qui modifient des indications sur leur entreprise pour leur apporter toutes les réponses qu'ils souhaitent. Je le redis, nous sommes au service des entreprises. Il doit néanmoins être corrigé dans son fonctionnement, ce qui sera fait dans les toutes prochaines semaines. Nous avons laissé à l'Inpi jusqu'au début du mois de mars, pas plus tard, pour que le site soit effectif, opérationnel, simple et d'accès direct pour tous les entrepreneurs. Monsieur le ministre, l'État a été prévenu très en amont des risques de dysfonctionnement. Dès l'automne 2022, des inquiétudes sur le caractère opérationnel du guichet unique se sont fait jour chez tous les professionnels qui accompagnent les entreprises : experts-comptables, avocats, notaires, etc.

Vous avez reconnu que le système nécessitait quelques optimisations- en effet ! -, mais aussi une protection efficace contre les cyberattaques. En catastrophe, un arrêté du 28 décembre 2022 a prévu une procédure de secours, de manière à assurer la continuité de service. C'est ce que font aujourd'hui les réseaux consulaires et Infogreffe. Ces derniers jouent les pompiers face au bug de ce lancement raté.

Sa famille avait pourtant signalé la situation au mois de septembre dernier. L'action de l'équipe pédagogique du collège n'a pas suffi. Une enquête diligentée par le parquet d'Épinal est en cours et déterminera les responsabilités de chacun.

J'avais déjà interpellé votre prédécesseur au sujet des messages haineux et violents présents sur les réseaux sociaux à l'encontre de collégiens. Dans sa réponse, le ministre avait rappelé l'importance du programme pHARe, dont l'ambition était l'avènement Monsieur le ministre, vous partagez cette ambition. Vous venez de le rappeler en réponse à l'intervention de notre collègue Mélanie Vogel. Encore faut-il que les dispositifs annoncés pour lutter contre l'homophobie soient efficaces. Au mois de novembre dernier, vous avez souligné les excellents résultats du programme pHARe.

en l'occurrence de harcèlement homophobe. Cette situation, comme vous l'indiquez, avait été signalée par les parents et prise en charge à l'automne par la communauté éducative du collège Louis-Armand de Golbey, dans votre département des Vosges. À l'évidence, cela n'a pas suffi. Une enquête est en cours, et nous aurons à en tirer les leçons. La loi Balanant, que vous avez votée, a fait un délit du harcèlement scolaire et a accentué la prise de conscience sur la gravité du phénomène. Vous l'avez dit, un élève sur dix est victime de harcèlement au cours de sa scolarité, avec des conséquences parfois catastrophiques.

de le généraliser, avec la création d'équipes d'élèves ambassadeurs et la formation de personnels référents. Nous avons aussi lancé une grande campagne de communication à propos des numéros 3020 et 3018. C'est d'ailleurs ce que préconisaient les sénatrices Mélot et Van Heghe dans leur rapport sur le harcèlement scolaire et sur le cyberharcèlement. Vous avez raison d'indiquer que le cyberharcèlement prolonge, en quelque sorte, les situations de harcèlement scolaire. Aussi, les plateformes de réseaux sociaux doivent faire plus

mais aussi d'autres métropoles, comme Nantes, sont victimes d'une véritable conquête de territoires par des trafiquants de drogue et par le crime organisé. Certains des habitants de ces quartiers se sont même mobilisés pour essayer d'empêcher l'installation du trafic et protéger leur famille en se relayant jour et nuit. Comment en sommes-nous arrivés là, monsieur le ministre ? Comment des quartiers autrefois tranquilles ont-ils pu se transformer en moins d'une génération en « Chicago-sur-Rhône » ou en « Bronx-sur-Loire » ? Quand des citoyens en viennent à devoir se protéger par eux-mêmes, c'est le début d'une lente déconstruction du processus de civilisation. L'État recule, les lois de la République s'effacent et la loi du plus fort s'impose à tous. Ce que subissent les habitants de ces quartiers, c'est la conséquence à la fois de l'explosion de la délinquance des mineurs, de l'effondrement de la chaîne pénale, de la surpopulation carcérale,

Aller beaucoup plus loin, c'est construire des prisons pour rétablir la chaîne pénale. Aller beaucoup plus loin, c'est condamner et incarcérer systématiquement les primodélinquants sur le chemin de la multirécidive. Aller beaucoup plus loin, c'est également en finir avec l'excuse de minorité. Aller beaucoup plus loin, c'est enfin, avant tout, enlever de l'esprit de certains consommateurs l'idée qu'acheter une barrette de cannabis, c'est comme acheter un tube de Doliprane

Républicain. Madame la Première ministre, depuis la présentation de votre projet de réforme des retraites, la colère gronde partout en France. Les Français sont très inquiets. Or vous avez décidé d'ignorer les partenaires sociaux. Votre projet n'est pas indispensable pour le moment ; il entraînera un recul social sans précédent. 70 % des Français refusent cette réforme injuste et injustifiée. Vous avez fait le choix d'humilier les syndicats. L'absence de concertation et de dialogue social s'apparente à un mépris volontaire. Demain, le pays s'arrêtera, compte tenu du front syndical uni qui appelle à la mobilisation contre votre projet. Après la crise sanitaire, la France a besoin de sérénité. Or vous avez fait le choix de la double peine,

Pourquoi choisissez-vous le chaos partout en France ? Pourquoi voulez-vous remettre au travail les plus pauvres, les plus fragiles et particulièrement les femmes ? La parole

Amélioré quant à la prise en compte des carrières longues, par une considération toute particulière apportée à ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, qui n'étaient jusqu'à présent pas plus protégés que ceux qui commençaient avant 20 ans, pour leur permettre un départ anticipé, là aussi,

la pension des retraités actuels qui ont les plus petits revenus après une carrière complète. Amélioré sur les retraites agricoles, amélioré aussi par la prise en compte des trimestres obtenus au titre de l'assurance vieillesse par les parents au foyer, de leur éligibilité au minimum de retraite, mais aussi à des départs anticipés pour carrière longue. Ce sont les concertations qui ont permis cela, madame la sénatrice ! Nous savons que, demain, il y aura une mobilisation ; je sais que, parmi les manifestants, beaucoup sont de bonne foi,

Pourquoi ce mépris à l'égard des syndicats ? Vous avez parlé de concertation. Mais pourquoi seront-ils demain dans la rue, unis ? Posez-vous les vraies questions ! Ce n'est pas parce qu'ils étaient à côté de vous que vous les avez entendus. Alors, faites l'effort nécessaire pour que les syndicats

dans le cadre de cette loi, mais il faut aussi assumer un discours clair devant les Français. Le bon prix, ce n'est pas le prix le plus bas : c'est le prix juste, celui qui permet de rémunérer le producteur. Celui-ci aime ses fruits. Je crois que c'est Félix Leclerc qui chantait : « Chaque pomme est une fleur qui a connu l'amour. » Il nous faut donc valoriser ces fruits

mais produire mieux : c'est tout le sens de la planification souhaitée par Mme la Première ministre. Ce sont des transitions que nous devons mener à l'échelle européenne, afin qu'elles ne pénalisent pas les producteurs français. Il convient aussi d'accompagner la filière en développant la recherche d'alternatives,

En arrivant à Beyrouth, l'odeur du fioul qui alimente les générateurs vous prend à la gorge. L'absence d'électricité m'a rappelé mon arrivée en Ukraine. En trois ans, la livre libanaise a perdu 90 % de sa valeur. L'inflation, sur un an, s'élève à 162 %. La crise bancaire a ruiné les Libanais. Le Liban connaît une aggravation de sa situation économique et sociale, qui a entraîné un exode massif, sans précédent, de la population active. Le blocage politique orchestré par le Hezbollah, qui a privé le Liban d'un président pendant plus de deux ans, se reproduit depuis le mois d'octobre. J'ai rencontré de nombreuses associations et des personnalités politiques de toutes tendances. J'ai pu apprécier le travail des équipes diplomatiques françaises, conduites par notre remarquable ambassadrice Anne Grillo, dans les domaines de la santé, de l'enseignement, des infrastructures ou encore Tous mes interlocuteurs louent l'action menée par la France pour aider les Libanais. Je vous le dis, madame la ministre, cette reconnaissance m'a procuré un grand sentiment de fierté pour la France et pour notre action collective.

Mes interlocuteurs m'ont demandé de relayer auprès de vous, madame la ministre, leur appel à tout faire pour que justice soit rendue. « Un crime impuni est un crime récompensé », m'a lancé un député. Des juges européens viennent d'arriver à Beyrouth, dont un juge français. Quels progrès pouvons-nous attendre de leur déplacement au Liban ? La parole

Nous le soutenons sur le plan politique, comme je l'ai fait au mois d'octobre dernier, comme vous l'avez fait récemment. Je le redis aujourd'hui : les responsables libanais doivent dépasser le blocage actuel et le Liban doit se doter d'un président ; un président doit être élu sans plus de délai Enfin, nous relayons l'aspiration du peuple libanais à la justice. Vous avez mentionné le déplacement de juges d'instruction français. Il s'agit d'une affaire judiciaire en cours ; il ne m'appartient donc pas de la commenter. la commenter. Quant à l'enquête relative à l'explosion survenue sur le port de Beyrouth le 4 août 2020, c'est une procédure distincte.

Pour être plus précise, elle doit être conduite à l'abri de toute interférence politique. La justice doit être rendue et les responsables doivent rendre des comptes. C'est donc bien volontiers que je réponds ainsi à votre appel, monsieur le

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ont été publiées.